danger, confrontée à de multiples crises et défis auxquels nous devons apporter des réponses adaptées, efficaces et pérennes. Le groupe Les Indépendants a choisi d'éclairer, par ce débat, ses difficultés, mais aussi ses atouts. Monsieur Monsieur le ministre, le moment est aujourd'hui opportun, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, de nombreux rapports récents sont venus étayer nos réflexions, comme celui de la Cour des comptes, publié en avril dernier, mais aussi celui de notre collègue députée Anne-Laure Cattelot, qui est

Aléas climatiques, développement de maladies ou encore présence de nuisibles, comme les scolytes et les chenilles processionnaires, sont autant de traces visibles d'une forêt victime de ces changements. La forêt est pourtant un levier essentiel pour lutter contre ce changement climatique et pour la préservation de nos ressources naturelles et de notre biodiversité. Nous devons aujourd'hui accompagner son adaptation et construire la forêt de demain. La stratégie de la transition écologique de la France doit passer par une gestion durable des forêts, par une politique renouvelée, stable et volontariste inscrite dans le long terme, long terme, couplée à des niveaux d'investissements et de recherches importants. La deuxième crise est d'ordre économique. Protéger notre forêt, c'est aussi l'entretenir, la gérer durablement et en valoriser les atouts. Notre filière forêt-bois constitue l'une des réponses principales : elle représente 440 000 emplois, soit 12,7 % de l'effectif industriel français, et pèse 60 milliards d'euros d'activités. Néanmoins, son déficit commercial de 6,8 milliards d'euros s'accroît de manière constante. Ces chiffres sont issus du rapport de la Cour des comptes,

La filière rencontre des problèmes dans ses approvisionnements, une fragilisation de la première transformation faute de débouchés et une concurrence des marchés étrangers sur la seconde ; d'où l'enjeu d'un travail approfondi en amont et en aval. La filière bois doit jouer un rôle majeur dans le secteur du bâtiment, notamment dans la rénovation. À titre de recommandations et à l'aune du plan de relance, nous devons la revaloriser et inciter davantage à l'utilisation du bois, véritable levier de la stratégie bas-carbone, dans la construction et le bâtiment. Nous sommes d'ailleurs en attente d'une réglementation La troisième crise que je souhaite évoquer est sociétale : la forêt est, pour beaucoup de Français, un lieu de loisirs, de découverte et de bien-être ; c'est aussi un milieu dans lequel l'équilibre sylvocynégétique est primordial. les déséquilibres parfois observés affectent la régénération des forêts. Un dialogue permanent entre les forestiers et les chasseurs est donc indispensable. Surtout, nous voyons se développer un courant de pensée selon lequel il faudrait protéger les arbres sans les exploiter. Mettre sous cloche la forêt reviendrait pourtant à ignorer que seule son exploitation durable permet sa régénération, en captant et en fixant le carbone. À la suite des auditions menées avec mon collègue Daniel Chasseing, je vous propose plusieurs pistes de réflexion.

forêts (ONF), ensuite, joue un rôle majeur. Il est pourtant indispensable de clarifier ses missions, de revoir son modèle économique, de lui donner les moyens de ses ambitions et de développer un dialogue plus systématique avec le local et la filière bois.

C'est l'occasion pour nous de réaffirmer le rôle essentiel des élus qui participent à la gestion des forêts communales et sont en première ligne dans la gestion de crise. Ils font le lien avec les propriétaires privés, avec l'ONF, avec la filière bois, avec les chasseurs, et doivent être les acteurs d'une territorialisation accrue de la stratégie forestière française. Ce point pose, par ailleurs, le problème de l'information et des données. En effet, le flux d'informations entre les acteurs est une part importante de la réussite d'une politique forestière cohérente. La lutte efficace contre les crises repose sur l'utilisation d'outils modernes, sur l'innovation, sur la recherche, sur le développement et sur des investissements importants. Enfin, venons-en au plan de relance, que je veux saluer, monsieur le ministre, même s'il m'inspire deux mises en garde. La première concerne la durée de deux ans prévue pour son déploiement. Le temps de la forêt est un temps long,

Ce plan de relance constitue véritablement un indispensable, qui devra être relayé par une politique de long terme. Je soutiens d'ailleurs, comme les acteurs de la filière, le projet de création d'un fonds sur trente ans pour l'avenir de la forêt, qui devrait être doté de 300 millions d'euros

et quel endroit est plus indiqué pour en débattre que cet hémicycle, placé sous le regard exigeant de Colbert, qui considérait la forêt comme un trésor qu'il faut soigneusement conserver ? Surtout, n'oublions jamais que la forêt est le fruit et l'oeuvre du travail des hommes

en soulignant le plaisir que j'éprouve à venir débattre ce matin avec vous de ce beau sujet qu'est la forêt française. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur Franck Menonville, les défis sont immenses ; la forêt est à la fois un patrimoine

La France est aussi un grand pays forestier, avec une forêt qui se cultive, qui est un élément très important de l'environnement dans lequel nous vivons et qui doit donc être protégée.

constitue pourtant également un atout majeur dans la lutte contre ces mêmes changements, car elle fait partie intégrante du cycle du carbone et constitue un réservoir de biodiversité, gage de résilience. Cependant, le morcellement de la propriété forestière rend sa gestion compliquée.

La recherche des biens non bâtis présumés sans maître est désormais de la compétence de l'État, mais les services de la direction des finances publiques sont souvent dans l'incapacité de la mettre en oeuvre complètement. On constate ainsi que les listes transmises aux mairies par l'intermédiaire des préfectures se limitent aux seules propriétés du domaine des propriétaires inconnus, ce qui est loin de recouvrir la notion de non-paiement des impôts fonciers pendant trois ans, prévue dans les textes. Monsieur le ministre, quelles solutions préconisez-vous pour faciliter la mise à jour des données cadastrales, aussi bien en termes de nature des cultures déclarées que pour la vérification des propriétaires dont les données cadastrales posent manifestement question ? La parole est

la disponibilité des informations relatives aux droits de propriété, ou plus exactement aux relevés de propriété. Vous insistez sur le fait que certaines de ces données ne sont pas suffisamment accessibles. C'est pourquoi j'ai introduit, dans le projet de loi d'accélération et

suggestion d'un meilleur suivi des remontées des commissions communales des impôts directs, du rappel de la nature de cultures déclarées sur les feuilles d'imposition, de celui de l'existence de surfaces en deçà du seuil de recouvrement des impôts fonciers,

dédiés à la forêt s'ouvre par un constat que nous partageons tous : nos forêts sont déjà durement touchées par le changement climatique, alors même qu'elles jouent un rôle essentiel dans la lutte contre ce même réchauffement climatique. On nous dit qu'il est impératif de financer l'amélioration, la diversification et le renouvellement des peuplements forestiers, afin de favoriser une meilleure résilience des écosystèmes forestiers, dans le respect d'une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt. Nous en sommes tous

Ainsi, depuis trois ans, les concours de recrutement de techniciens forestiers fonctionnaires sont bloqués et les postes de gardes forestiers sont affectés massivement à des contractuels. Enfin, le Gouvernement a annoncé un plan de soutien à la filière bois, mais il ne prévoit aucune augmentation du budget de l'ONF, pourtant en déficit structurel depuis plusieurs années. La conséquence de ces politiques est un affaiblissement de la protection des forêts. Dès lors, monsieur le ministre, quand allez-vous décider de mettre un terme à cette spirale de destruction d'un outil si précieux, indispensable pour assurer la durabilité de nos forêts ? La parole est à

cela me paraissait absolument nécessaire. Sur les trois points que vous évoquez, les financements que nous devons octroyer à l'ONF sont importants et doivent prendre en compte, effectivement, la situation financière actuelle de l'Office, que vous avez rappelée. Il y a,

pour lesquels je considère la forêt comme une solution : réchauffement climatique, menaces sur la ressource en eau, glissements de terrain, érosion de la biodiversité, biodiversité, demande de nature de nos concitoyens. La forêt peut assumer de nombreuses fonctions, si tant est qu'elle fasse l'objet d'une gestion

est ambitionné, ainsi qu'un renforcement des dispositifs de soutien aux entreprises de la filière bois. Monsieur le ministre, cette démarche va dans le bon sens,

quelles seront les modalités du volet forêt de la relance ? Le développement forestier ne se décrète pas : il se construit de manière volontaire et concertée avec les acteurs locaux, autour, surtout, d'un projet commun qui profitera à nos territoires ! La parole

Les forestiers privés sont également touchés : les rendements s'effondrent sous l'effet d'une chute des cours, et les marchés régionaux sont saturés. À long terme, nous sommes face à un problème de pérennité de nos couverts forestiers.

le réchauffement climatique est jugé par la majorité de l'opinion comme une certitude absolue, la forêt étant une affaire de long terme, nous avons le devoir absolu, face à un horizon de

Le dérèglement climatique, l'infestation par les hannetons et les dégradations causées par le grand gibier : en dix ans, les gestionnaires, dont évidemment l'ONF, ont pu identifier les causes majeures des problèmes de la forêt de Chantilly. Une mobilisation importante s'est déployée pour agir et conserver une forêt vivante. Elle a permis de mettre autour de la table tous les acteurs : la population, les scientifiques, les associations environnementales, les chasseurs et les élus. Ainsi, les problèmes ont pu être identifiés, et les solutions dégagées. Les solutions, nombreuses, s'inscrivent dans un schéma national : le reboisement, l'inclusion des chasseurs dans les discussions de régénération de la forêt, l'adaptation de la forêt par la recherche et le développement d'actions en faveur de la filière bois, dans le respect de ses particularités, afin d'assurer son avenir. Pour établir un cadre et organiser au mieux cette action, l'idée a émergé de créer un groupe d'intérêt public. Loin d'être un comité Théodule, ce GIP met tout le monde autour de la table pour travailler à l'organisation et l'aménagement d'une gestion durable et adaptée au domaine forestier, avec un objectif principal : trouver des solutions face aux dangers qui guettent la forêt. Je souhaitais attirer l'attention sur le combat mené pour la forêt de Chantilly, parce qu'il y a urgence ! Monsieur le ministre, cette pratique volontariste et la création de ce GIP ne pourraient-elles pas être dupliquées, en tenant compte des spécificités de chaque situation

voilà quelques jours, l'Anses a été très claire sur l'utilisation du glyphosate en forêt,

la forêt couvre 8 millions d'hectares, soit 96 % du territoire. Or l'État a confié 6 millions d'hectares de son domaine privé au seul Office national des forêts. en Guyane, et nulle part ailleurs, d'un rôle de conservateur gestionnaire, mais aussi d'opérateur, ce qui fait de ses agents des juges et parties dans bon nombre de dossiers. En 2015, la délégation sénatoriale aux outre-mer a émis trente propositions pour « mettre un terme à une gestion jalouse et stérile du domaine public et privé de l'État en outre-mer ». Elle a proposé une nouvelle architecture propre à la Guyane, destinée à libérer du foncier d'État au service du développement local. Il s'agirait notamment d'accélérer les procédures de cession de terrains du domaine privé, de repousser vers l'intérieur des terres les limites du domaine forestier permanent et de transférer le foncier libéré à la collectivité unique de Guyane, charge à elle de le rétrocéder aux communes et aux acteurs économiques. Monsieur le ministre, l'exploitation du bois et des produits de la forêt constitue une filière d'avenir pour la Guyane, mais l'accès à la ressource reste problématique, car l'ONF demeure l'unique fournisseur de bois pour les professionnels de la première transformation. L'État semble réticent à laisser une partie de la maîtrise foncière à la collectivité territoriale de Guyane, qui, en cas de rétrocession, disposerait d'un levier permettant de mettre en oeuvre une véritable politique de développement économique. Pourtant, après les événements de 2017, l'État s'était engagé à transférer 250 000 hectares à la collectivité territoriale de Guyane. Malheureusement, ce transfert n'a toujours pas eu lieu, alors qu'il pourrait éviter certaines crispations au sein de la population sur des problématiques telles que la chasse

d'approvisionner les industries de la filière bois, et surtout d'accroître la capacité des forêts à capter du carbone, lesquelles contribueront ainsi au respect des engagements climatiques de la France. Le Gouvernement a rappelé à juste titre que la filière bois permettait de compenser environ 20 % des émissions françaises de CO2 et qu'elle jouait ainsi un rôle majeur en matière d'atténuation du changement climatique. Pour autant, ce rôle repose sur la résilience des forêts, notamment sur leur capacité à s'adapter à ce changement. Vous avez donc prévu un grand plan de reboisement allouant 150 millions d'euros à la plantation de 45 000 hectares de forêt afin d'augmenter les surfaces plantées, de régénérer les surfaces existantes et de reconstituer celles qui ont dépéri, notamment en raison des attaques de scolytes. J'attire néanmoins votre attention sur le fait que l'attribution de ces crédits à la plantation ne semble à ce stade ni conditionnée à une certification de gestion durable Or dans le contexte actuel, nous observons de fortes interrogations sociétales sur la gestion forestière. Il me semble particulièrement important de donner à nos concitoyens la certitude que l'État a tout mis en oeuvre pour s'assurer que le propriétaire forestier qui bénéficiera de cette importante aide publique au reboisement l'utilisera en respectant des critères de durabilité inscrits dans la démarche de certification forestière. Pour ce faire, le Gouvernement pourrait conditionner l'attribution des aides publiques à l'adhésion à une certification de gestion durable des forêts,

accompagné d'un renfort de sapeurs-pompiers hexagonaux. Cette tragédie vient rappeler l'importance de la forêt pour cette île tropicale montagneuse de l'océan Indien. La Réunion est en effet l'un des trente-cinq de biodiversité terrestre mondiale. Sa richesse patrimoniale et ses taux d'endémisme records sont reconnus à l'échelon planétaire. Depuis 2010, l'inscription des pitons, cirques et remparts au patrimoine mondial de l'Unesco est pour nous une fierté. de cette distinction ne pourra se faire sans le concours de l'Office national des forêts, qui gère plus de 90 % du domaine forestier de l'île. Monsieur le ministre, l'action de l'ONF sur notre territoire est reconnue de tous, notamment en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de prévention des risques naturels, mais aussi d'entretien des 850 kilomètres de sentiers, des 365 aires d'accueil du public en forêt, des 609 kilomètres de routes et de pistes forestières, des 276 kilomètres de pistes de VTT et des 158 kilomètres de pistes équestres, qui sont dégradés après chaque saison cyclonique et représentent des enjeux importants pour le tourisme. Le faible niveau de production forestière à l'échelon local, le surcoût lié à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco et les autres activités hors du régime forestier, financées partiellement ou non financées, expliquent le déficit structurel de l'ONF de La Réunion. Or la réduction des moyens humains et financiers de l'ONF sur l'île semble engagée. Le projet de contrat État-ONF pour la période 2021-2025 nous inquiète fortement, car il ne fait pas mention de La Réunion.

au marché. Elle a une fonction économique irremplaçable, mais aussi une fonction environnementale pour le maintien de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique- elle est un formidable piège à carbone. Enfin, elle a une fonction de protection contre les risques naturels, notamment

la forêt méditerranéenne s'étend sur tout le sud de la France, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'Occitanie, de la Drôme à la Corse. Elle représente un tiers de la forêt française. Longtemps prisé par les constructeurs, le pin d'Alep a été abandonné au XX siècle au profit d'alliages de nouveaux métaux, et toute l'économie sylvicole l'entourant a pratiquement disparu. L'industrie revenant vers des matériaux naturels, ce résineux résistant présente de nouveaux atouts. Pourtant, sa production est considérablement freinée, d'une part parce que sa normalisation comme bois d'oeuvre n'est intervenue que très récemment, part parce que la relance d'une économie dédiée requiert des investissements importants sur le moyen terme. Les acteurs publics locaux sont prêts à investir pour soutenir des partenaires publics et privés, mais la limite européenne des 40 % d'aides publiques à l'investissement bloque les projets de relance, car la forêt méditerranéenne est peu productive comparée à d'autres forêts nationales. L'actuelle renégociation de la politique agricole commune (PAC) est le moment opportun pour défendre la spécificité de cette forêt et le bien-fondé d'une action publique soutenue.

C'est un engagement environnemental fort pour les générations futures. La production de bois d'oeuvre est la seule solution pour capter du carbone de façon permanente. Se contenter de couper la forêt pour produire de la biomasse ne ferait que décaler le relâchement des émissions de CO2 d'un demi-siècle. de l'argument écologique, l'investissement dans la forêt méditerranéenne est une stratégie ambitieuse pour développer l'économie locale, créer des emplois et des richesses dans des territoires ruraux. l'État semble enfin avoir pris la mesure de la nécessité de faire évoluer l'encadrement des aides publiques à l'investissement en forêt. C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de ne pas oublier la forêt méditerranéenne et de lui permettre de bénéficier d'une hausse des taux d'aide publique à l'investissement forestier.

nette augmentation du bois dépérissant, engorgement du marché du bois et chute des prix. Nos repères s'écroulent, et tous les indices confirment qu'un scénario de crise se met inexorablement en place. L'heure est venue de réinventer la forêt, de donner l'envie, mais aussi les moyens aux propriétaires forestiers de reboiser leurs forêts sinistrées. Aujourd'hui, l'intérêt financier d'un boisement est difficile à démontrer. Or il est indispensable de maintenir notre patrimoine forestier.

l'attribution des aides forestière nécessite de constituer des dossiers complexes. Si cette procédure est bien adaptée aux boisements importants, elle ne l'est pas pour les petites plantations. Dans le contexte du réchauffement climatique, il est intéressant de constituer des îlots d'avenir et des enrichissements de régénération naturelle. Jadis, dans le cadre du Fonds forestier national, il était possible d'obtenir des bons de subvention pour de petits reboisements. Par le biais d'un formulaire simple, le propriétaire adressait sa demande à l'administration, et il pouvait retirer ses plans gratuitement auprès d'une pépinière agréée.

Nos forêts sont singulièrement concernées par cette invasion qui fait des ravages. Or il n'existe pas de remède contre les scolytes. Les communes forestières vont donc être contraintes de revoir totalement le modèle de développement de leur forêt. Le réchauffement climatique entraîne une surpopulation de ces insectes, de plus en plus d'arbres résineux sont touchés. Parallèlement, la sécheresse sévit dans les plantations de feuillus, provoquant leur dépérissement.

: premièrement, en augmentant la dotation de solidarité rurale pour les communes forestières afin de compenser le manque à gagner de ces trois années ; deuxièmement, en aidant de manière significative les communes à repeupler leurs forêts

et la régulation des risques naturels. Ces enjeux environnementaux représentent une opportunité dont il faut nous saisir. La forêt française est privée à 74 %. Encourager fiscalement la gestion de la forêt privée aura un effet direct sur l'atteinte des objectifs environnementaux. tel dispositif d'encouragement sera dérisoire par rapport aux bénéfices globaux en matière de changement climatique. La loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001

simple, est également très opérationnel pour accompagner l'investissement forestier. Toutefois, son manque de lisibilité et ses modifications successives ont rendu son utilisation complexe. Au regard des enjeux climatiques et économiques pour la forêt française, il est nécessaire que l'État favorise l'investissement et la gestion durable des forêts privées, non seulement en reconduisant la mesure, mais en l'améliorant fortement. Monsieur le ministre, le Gouvernement a accepté de prolonger de deux ans ce dispositif d'encouragement fiscal. Or, dans

sur le long terme. Nous partageons tous le constat que l'inaction serait dévastatrice pour notre environnement, notre économie et notre société. Un tiers de notre territoire métropolitain est occupé par la forêt.

la sauvegarde de notre biodiversité et de nos ressources naturelles. Nous devons la protéger, l'aider à s'adapter et à se régénérer pour faire face aux défis auxquels elle est confrontée.

les difficultés économiques auxquelles elle est confrontée. Je m'attarderai sur le secteur du bâtiment. En effet, le bois a des qualités et une performance thermique dont nous aurions tort de nous passer. Il peut être utilisé dans la rénovation, mais aussi dans le neuf. La construction d'une maison en bois réduit de 55 % les émissions de CO2, ce qui est un atout dans un secteur qui représente 40 % des émissions mondiales.

des conséquences positives sur la création d'emplois et la valorisation de la filière. Cependant, il faut surtout inciter les propriétaires à se restructurer, comme l'ont suggéré plusieurs de mes collègues. Monsieur le ministre, un travail

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il y avait autrefois dans les villages celui qu'on appelait l'idiot du village. Aujourd'hui, les idiots du village global sont sur internet. Ils croient que la terre est plate ou que la lune est habitée parce qu'il y a de la lumière la nuit. Ils sont complotistes, harceleurs, racistes, haineux, radicalisés ou délirants. Cela n'aurait pas beaucoup d'importance si les réseaux sociaux ne leur permettaient de se reconnaître, de se rassembler et de se réunir. On s'aperçoit alors qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le croyait. Staline demandait : « Le pape, combien de divisions » ? L'armée des idiots du village en a beaucoup. Pourquoi s'en préoccuper ? Après tout, peut-être vaut-il mieux laisser délirer entre eux ceux qui croient que Bill Gates veut tuer 15 % de l'humanité avec un vaccin contre la covid ... Mais les choses ont changé depuis que Facebook, au lendemain de l'élection américaine de 2016, a modifié ses algorithmes qui avaient permis aux de peser sur le résultat du vote. Dégrader la promotion des pages au profit des groupes partait d'une idée intéressante, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions une grande partie du contenu des fils d'actualité proviennent aujourd'hui des groupes et de leurs centaines de liens, de vidéos et de commentaires indignés. Les plateformes sont désormais remplies de bataillons soudés à l'intérieur par leurs certitudes et leurs indignations, et à l'extérieur par le combat contre ceux qui ne pensent pas comme eux. des groupes sur Facebook, des combattants sur Twitter, le tout exacerbé par YouTube, une bonne partie de l'écosystème des réseaux dits « sociaux » ressemble chaque jour un peu plus à des gangs rivaux s'agressant dans des quartiers mal famés. « Nul ne ment autant qu'un homme indigné », écrivait Nietzsche. Et le mensonge est devenu généralisé, favorisé par l'anonymat et la certitude de l'impunité. Le mensonge, mais aussi l'injure, la haine, le sexisme, le racisme, l'homophobie, les menaces, la violence, la propagande terroriste tout un pan de l'internet est devenu un dépotoir. Ce qui est grave, ce sont les conséquences, celles qui s'exercent sur la vie des victimes du harcèlement, du, des dénonciations, des menaces de mort. Beaucoup ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils n'ont pas été victimes personnellement des tombereaux de boue déversés quotidiennement. Ils n'ont pas été forcés de fermer leurs comptes en ligne, de changer d'école ou de ville, leur réputation n'a Ils ne sont pas obligés de vivre chaque jour sous protection policière, comme Sonia Mabrouk, comme Zineb El Rhazoui et tant d'autres, victimes de fatwas sur internet. Mais le phénomène a pris tant d'ampleur que personne ne peut plus fermer les yeux. L'affaire Mila, médiatisée dans tous ses détails et dans toute son horreur,

Il est urgent de se donner des lois enfin efficaces contre la haine en ligne. Ce ne sera pas facile en raison de l'obstruction des plateformes, qui luttent pied à pied contre les régulations, parce que c'est leur même qui est en cause.

la polarisation de notre société fait partie du modèle commercial des réseaux sociaux. » Bien sûr, les plateformes ne peuvent pas avouer la raison de leur passivité : le pognon Alors, leurs milliers d'avocats et de lobbyistes partent à l'assaut des gouvernements, des parlements et des opinions publiques avec un argument massue : la liberté d'expression. Et malheureusement, cela marche souvent, comme on l'a vu lors du débat sur la loi Avia. Celle-ci ne prévoyait pas une privatisation de la censure, elle ne visait pas à confier aux plateformes ce qui relève du juge. C'est aujourd'hui que la censure existe, et elle est toute-puissante. La censure, ce sont les milliers d'internautes qui n'osent plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui ont résilié leur abonnement pour ne plus s'exposer aux attaques racistes, antisémites, homophobes et sexistes, menées sous forme de raids en bandes organisées, ou de « fermes de trolls » submergeant les pages individuelles. C'est là qu'est le scandale, c'est là qu'est la censure Comment peut-on soutenir que le retrait des contenus haineux porte atteinte à la liberté d'expression ? La liberté d'expression, ce n'est pas la diffusion de la haine, de la violence, des appels au meurtre ou au viol ; ce n'est pas non plus empêcher les autres de s'exprimer par des attaques massives ou des menaces. En confondant ces délits avec la liberté d'expression, ce ne sont pas les victimes que l'on défend, ce sont les agresseurs. Comment comprendre que l'on n'impose pas aux plateformes ce que l'on impose à la presse depuis 1881 : l'interdiction de livrer des contenus haineux, diffamatoires ou injurieux ? La presse s'y conforme évidemment, et personne n'a jamais dit qu'on lui confiait le rôle de juge. Et bien sûr que plateformes et presse ont les mêmes responsabilités.

Pourquoi cette évidence est-elle si difficile à faire comprendre ? Le projet de loi annoncé hier par le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux est bienvenu, mais, d'une part, il ne traite qu'un aspect du problème

pour une modération effective, réelle et efficace. « C'est très cher », nous disent-elles en gémissant. De tels propos sont indécents de la part des sociétés les plus riches du monde. Le combat sera difficile puisqu'il s'agit d'une collision frontale avec le actuel des réseaux, mais il y va de la lutte contre les incendiaires du web, de la sécurité des victimes et,, de la stabilité de nos démocraties. Pour ceux qui penseraient que j'exagère, je citerai Barack Obama, qui a déclaré lors d'un entretien donné il y a quelques jours à : « L'internet et les réseaux sociaux sont devenus une des principales menaces contre la démocratie. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur le gouvernement français pour convaincre l'Europe de ne pas se satisfaire de demi-mesures. Jean Castex nous l'a promis ici même il y a quelques jours, et vous l'avez dit sur votre blog, monsieur le secrétaire

si l'on n'est pas capable de réguler efficacement internet et de protéger nos concitoyens, ces derniers finiront par opter pour des solutions plus radicales.

-qui viennent chercher le contact et le réconfort lors de parties de jeux vidéo en ligne. Au contraire, faut-il être permissif, comme les éditeurs qui laissent tout passer et prospérer des pseudonymes nazis et des insultes raciales ?

Si, pour une partie d'entre eux, ils ne fraudent pas dans le métro, c'est parce qu'ils ont peur de se faire attraper par les contrôleurs. Aujourd'hui, cette peur n'existe pas sur internet : vous savez que vous n'avez quasiment aucun risque de vous faire attraper.

nos référentiels institutionnels ont du mal à passer le cap de ces plateformes et que l'on ne parle pas la même langue. L'éducation de la jeunesse, les pratiques, les régulations, la dimension pédagogique

il faut lutter contre la haine sur internet, de la même manière qu'on lutte contre la haine dans l'espace public physique. C'est d'ailleurs ce que nous avons tenté de faire dans la proposition de loi Avia, nous avons eu l'occasion de débattre avec vous, monsieur le secrétaire d'État, et dont j'étais le rapporteur ici au Sénat. Cependant, et vous en conviendrez, je l'espère, ce n'est pas tant aux plateformes qu'il faut s'en prendre qu'aux auteurs de propos haineux, à ceux qui sont à la source des discours de haine. Or, un an après l'examen de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, les moyens ne sont à l'évidence pas là. Comment comprendre, monsieur le secrétaire d'État, qu'aujourd'hui encore, seul un nombre extrêmement réduit de services d'enquête et de poursuite,

comment imaginer pouvoir lutter efficacement contre les contenus antisémites et homophobes ? Nous avions fait un certain nombre de propositions constructives, au premier rang desquelles une meilleure régulation des plateformes par l'instauration d'obligations de moyens, sous la supervision d'un régulateur. Quoi qu'il en soit, le Conseil constitutionnel a eu raison de la loi de Mme Avia. Au-delà de l'incrimination pénale qui est annoncée, monsieur le secrétaire d'État, que comptez-vous proposer dans le futur projet de loi de lutte contre le séparatisme pour renforcer la lutte contre la haine en ligne ? monsieur le ministre,

Monsieur le secrétaire d'État, comme il y a un bon usage du monde, il doit y avoir un bon usage de la liberté d'expression en démocratie, tant celle-ci nous est précieuse et tant nous y sommes attachés.

Si les réseaux sociaux sont des espaces propices à l'exercice de la liberté d'expression, ils ne sont heureusement pas les seuls. Ces plateformes sont, je le rappelle, des espaces régis par des acteurs privés qui ont, comme le disait le président Malhuret, des, qui font des usagers leurs produits et qui ont leur propre vision de la liberté d'expression. Je vous rappelle que celle-ci n'est pas nécessairement la même que celle de la loi, comme l'a illustré la publication du tableau, qui a été censurée par Facebook,

ne serait-il pas judicieux, à titre préventif et à des fins d'autorégulation, de ne permettre aux usagers d'accéder aux réseaux qu'une fois leur identité enregistrée, d'une part, et d'ajouter aux sanctions déjà prévues par la loi des interdictions temporaires d'accéder à ces réseaux,

à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Sans empêcher le pseudonymat, une telle levée de l'anonymat, couplée à ce type de sanctions, pourrait avoir selon nous un fort pouvoir pédagogique : elle permettrait de responsabiliser les individus, qui ne doivent plus impunément se comporter comme des chauffards sur ces autoroutes de l'information.

sur notre capacité à juguler ces vagues massives de haine qui s'expriment en ligne, avec un sentiment d'impunité insupportable. Comment est-on passé de l'internet émancipateur des origines à ces réseaux d'oppression organisée et au harcèlement de masse ? On doit s'interroger sur les mécanismes principalement économiques qui ont conduit au succès des discours haineux sur certaines plateformes.

Si la loi doit être la même pour sanctionner l'expression des propos haineux en ligne ou hors ligne, on doit nécessairement s'interroger sur la massification de ce type de propos sur les grandes plateformes commerciales et sur la réponse judiciaire qu'il convient d'y apporter, tant leur nombre est démultiplié. d'une masse croissante d'utilisateurs et d'utilisatrices, se livrent à une compétition économique autour de la captation de notre attention. Pour cela, elles emploient chacune des mécaniques commerciales qui privilégient la diffusion des publications suscitant le plus d'engagement et enferment les utilisateurs dans des réseaux de plus en plus polarisés. Les propagateurs de haine l'ont bien compris et s'appuient sur ces mécaniques pour diffuser leurs messages. Face à ces plateformes, qui comptent des milliards d'utilisateurs et dont les modèles économiques valorisent les discours choquants, l'enjeu pour nos sociétés de liberté est d'être capables à la fois de réguler fortement ces mécaniques économiques favorisant les campagnes haineuses et de nous donner les moyens de briser le sentiment d'impunité. L'accélération des phénomènes de viralité, encouragés par les algorithmes des grandes plateformes,

fait que les gens ne comprennent pas bien ce qui se passe sur internet, ne serait-ce que parce qu'un Français sur six n'utilise jamais un ordinateur et qu'un sur trois manque de compétences de base. Certes, il faut apprendre aux gens à déclarer leurs impôts en ligne, à garder le contact avec leurs proches sur un réseau social, à rédiger un.

L'intitulé de ce débat est révélateur à lui seul de la complexité du sujet. Nous nous accorderons tous sur l'idée que notre pacte social ne peut souffrir d'atteintes sur internet, lesquelles seraient tolérées au motif qu'elles sont virtuelles. Les conditions dans lesquelles vit aujourd'hui l'adolescente Mila, que nous devons tous entourer de notre protection, montrent bien, si cela était encore nécessaire, que la menace n'est pas seulement en puissance, pour reprendre le sens étymologique du mot « virtuel ». Les conséquences de la haine en ligne sur les vies de nos concitoyens sont concrètes et souvent destructrices. Partant de ce constat nécessaire, la tâche n'est pas aisée, justement parce qu'internet a ses mécanismes propres, qui ne sont pas réductibles aux échanges hors ligne et qui sont assortis de régimes juridiques complexes. Je pense notamment à la dichotomie, qui pose parfois question, entre éditeurs de contenus et hébergeurs, ces derniers répondant d'une responsabilité allégée. Ainsi l'enjeu est non pas tant d'appliquer les mêmes lois en ligne et hors ligne que de bien adapter notre législation à l'espace numérique, afin d'y garantir le respect de nos droits et la même protection pour tous

Plusieurs pistes ont pu être utilement évoquées sur le sujet au cours des dernières semaines. Je pense au renforcement de la diligence et des obligations de moyens des plateformes, ou encore à la transparence sur la modération des contenus, s'agissant plus particulièrement des algorithmes

je vous remercie

rôle croissant des réseaux sociaux et multiplication des, affaiblissement du lien collectif au profit d'une forme d'individualisme, voire de communautarisme. Ces défis concernent également l'Europe, qui subit, elle aussi, une perte collective de repères et de confiance, sapant les fondements démocratiques. En France, la même démagogie, le même complotisme et le même cynisme se répandent. Les réseaux sociaux en sont un formidable vecteur, avec leur lot toujours plus important de menaces et d'intimidations, lancées derrière un écran, sous couvert d'anonymat et avec un fort sentiment d'impunité. C'est ainsi que l'on retrouve jetés en pâture tous les amalgames possibles, sans le moindre discernement et le moindre contrôle. Les petits paysans sont comparés à des assassins qui empoisonnent, les migrants à des terroristes, et toutes les règles élémentaires sont systématiquement remises en cause. Le projet de loi confortant les principes républicains, présenté cette semaine, contient certaines dispositions relatives à la haine en ligne permettant d'élargir le champ d'action de la justice. Mais aucune loi n'empêchera jamais ces discussions de comptoir sur internet, qui peuvent mener à la violence, sans le filtre de la conversation et du débat éclairé. Seule l'éducation en limitera les effets. C'est pourquoi l'investissement de l'État dans la lutte contre l'illectronisme pourrait être l'occasion de renforcer la sensibilisation des plus jeunes à ces sujets, conformément aux recommandations de la mission d'information créée, à la demande Cela ne doit surtout pas nous faire oublier la responsabilité des réseaux sociaux et leur modération à géométrie très variable. Comment l'État peut-il agir pour que ces réseaux sociaux et les forums renforcent l'efficacité de leur modération ? ? Entend-il investir davantage dans l'intelligence artificielle pour une modération plus opérationnelle dans ce domaine, mais aussi pour repérer efficacement les auteurs de discours appelant une

Aujourd'hui, les développeurs et les spécialistes de l'intelligence artificielle des GAFA sont les meilleurs du monde et sont payés plusieurs millions d'euros par an. La compétence disponible au sein de l'État pour ouvrir ou contrôler les boîtes noires,

avons commencé à travailler sur ce sujet en créant le pôle d'expertise de la régulation numérique. Cette structure rassemble des spécialistes du et de l'intelligence artificielle

sur le terrain et en ligne.

Le Gouvernement travaillerait d'ailleurs sur un dispositif juridique de lutte contre la haine sur les réseaux sociaux, à la suite de la censure de l'essentiel des dispositions de la loi Avia par le Conseil constitutionnel. Nous considérons, pour notre part, que la loi ne peut pas être la même hors ligne et en ligne. Même si, de toute évidence, ses grands principes doivent partout prévaloir, elle doit être adaptée à ce support immatériel et protéiforme.

Bien sûr, internet n'est autre que la continuité du monde qui nous entoure. Les propos haineux ne naissent pas sur internet, mais les géants de la toile, par leur modèle économique, favorisent leur diffusion et leur viralité. Il est donc nécessaire de penser un autre modèle d'interaction pour s'extirper de ces plateformes toutes-puissantes.

Nous sommes convaincus que cela permettrait d'enrayer la diffusion de contenus haineux sur internet, ou tout au moins de les limiter fortement. Monsieur le secrétaire d'État, quelle est votre position sur ce sujet précis et que pensez-vous de cette proposition ? La parole

Morin-Desailly. Oui, en ligne et hors ligne, la réponse doit être la même. Encore faut-il que la justice ait les moyens de lutter contre ce qui relève de la cybercriminalité. Aujourd'hui, elle trois personnes pour cela. Cela étant, force est de constater l'inefficacité des dispositions issues de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information ou encore de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, texte copieusement censuré par le Conseil constitutionnel. Je n'en suis pas étonnée, le Sénat avait indiqué à plusieurs reprises que les dispositions proposées, faisaient le jeu des plateformes et, au pire, portaient atteinte à nos libertés fondamentales. Au-delà du bon vouloir des plateformes, internet exige une véritable régulation et, donc, une réponse globale, structurelle et européenne. Cambridge Analytica nous avait déjà avertis sur la perméabilité et la vulnérabilité des démocraties face aux Gafam. La multiplication des appels à la haine et surtout leur viralité nous imposent d'ouvrir les yeux sur leurs conséquences dramatiques pour notre sécurité nationale l'influence des algorithmes utilisés par YouTube ou Facebook sur la radicalisation en ligne n'est plus un secret, le modèle de l'économie de l'attention favorisant toujours plus les contenus violents, extrémistes et haineux. Dans son ouvrage, l'universitaire américaine Shoshana Zuboff dénonce le détournement de nos données personnelles à des fins de manipulation des comportements et de radicalisation des opinions publiques. Avec le, la Commission européenne a enfin prévu la révision de la directive e-commerce, révision en passe d'aboutir, je l'espère, à de véritables

! Ce qu'il faudrait, c'est créer des consensus contre la haine et contre tous ceux qui en font commerce. Et pour créer des consensus, il faut arrêter d'utiliser

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, internet est un formidable vecteur de communication, mais le rôle des réseaux sociaux, en particulier, fait débat : on y côtoie le meilleur comme le pire. Il faut se réjouir quand ils permettent de donner corps à des initiatives solidaires en revanche, il faut les dénoncer et agir lorsqu'ils sont utilisés pour dégrader l'image d'un élu, d'un journaliste ou bien d'une personnalité, ou encore pour véhiculer certaines idéologies ou les thèses les plus abjectes. Il ne s'agit- hélas ! -que de la partie émergée de l'iceberg. Tous les jours, des utilisateurs sont victimes d'un harcèlement devenu ordinaire qui expose leur vie, leurs photos, leur identité, leur adresse ou leur profession à la connaissance de tous. L'ignominie du meurtre de Samuel Paty doit nous faire réfléchir sur les dérives inacceptables d'internet et sur la nécessité de le réguler. Des solutions existent, mais une prise de conscience et une action collective à l'échelle européenne sont nécessaires, comme le souligne très justement mon ami Geoffroy Didier, député au Parlement européen. Cela peut consister à imposer aux futurs utilisateurs des réseaux sociaux la présentation du d'une pièce d'identité lors de la création du compte. La fin de l'anonymat complet sur internet ne doit pas être un sujet tabou, et cela n'a rien à voir avec une quelconque remise en cause du droit à la vie privée. Pourquoi ne pas contraindre également chaque réseau social à afficher sur sa page d'accueil un lien vers le site gouvernemental de pré-plainte en ligne, afin de permettre aux victimes de harcèlement, d'insultes ou de menaces d'exercer pleinement leurs droits ? Simplifions les démarches pour une efficacité accrue contre les violences illégitimes Enfin, il serait judicieux de faire évoluer la nature juridique des plateformes, qui ne doivent plus s'abriter derrière leur statut d'hébergeur pour s'exonérer de toute responsabilité lorsqu'elles assurent la diffusion de messages contraires aux valeurs et à la dignité humaine. Utilisons le levier du droit ! Ma question est la suivante, monsieur le secrétaire d'État : êtes-vous prêt à vous engager sur ces mesures de bon sens, qui ne restreignent pas la liberté d'expression, mais permettent d'en limiter les excès ? Êtes-vous prêt à mener ce combat avec nos partenaires européens ? Notre réponse n'a que trop tardé ; il nous faut protéger les victimes et mettre un terme avec la plus grande énergie aux dérives d'internet. Je remercie le président Malhuret d'avoir suscité ce débat.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi confortant les principes républicains va donc nous permettre de reprendre la loi Avia. d'abord, je voudrais exprimer un point d'incompréhension ou d'incohérence. Sur la haine en ligne, vous voulez agir sans attendre l'Europe, ou, plus précisément, dans l'attente de sa première copie, qui sera présentée par la Commission européenne le 9 décembre prochain. Mais, sur l'encadrement économique, qui est au coeur du modèle numérique, vous vous êtes opposé aux propositions du Sénat. Pouvez-vous nous expliquer cette volte-face doctrinale ? S'agissant du sujet qui nous occupe aujourd'hui, je m'interroge sur plusieurs points quant à la méthode suivie. Je comprends que vous souhaitez réintroduire, par amendements, les dispositions de la loi Avia dans un second temps. Pourquoi en passer par cette voie, alors qu'un réexamen par le Conseil d'État n'aurait sans doute pas fait de mal, au regard de l'histoire légistique problématique de ce texte ? Deuxième question : vous engagez-vous à reprendre les avancées votées par le Sénat lors de l'examen de la loi ? Notre Haute Assemblée avait attiré l'attention sur le fait qu'il n'y avait pas que l'outil du retrait pour lutter contre les contenus haineux et qu'il convenait que les plateformes proportionnent leur action aux risques encourus. Le Sénat avait notamment insisté, à juste titre, sur le fait que la réduction de la visibilité d'un contenu et de sa viralité peut être un moyen tout aussi pertinent et davantage proportionné. Ces avancées figureront-elles dans votre projet ? Dernière question : le texte européen sur le retrait de contenus terroristes en une heure semble enlisé. Pensez-vous légiférer également sur ce point à cette occasion ? La parole

des forces de l'ordre, qu'ils soient fonctionnaires de police nationale, gendarmes ou encore policiers municipaux. Ces appels à la haine ont souvent comme support des images de ces agents filmés dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Nombre d'entre elles sont diffusées sur les réseaux sociaux, rendant ces agents facilement identifiables, les transformant, ainsi que leurs familles, en cibles potentielles. Ils ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une opération de police : la liberté de l'information, qu'elle soit le fait de la presse ou d'un particulier, prime le respect du droit à l'image ou à la vie privée. Ils ne peuvent donc s'opposer à l'enregistrement de leur image et, surtout, à son éventuelle diffusion malveillante. Aucune contrainte légale ne permet aux policiers de demander le floutage de leur visage avant la diffusion des images afin de garantir leur anonymat, floutage gage de leur efficacité, mais aussi de leur sécurité.

Monsieur le secrétaire d'État, si les divergences d'opinions sont nécessaires pour faire vivre notre démocratie, les discours de haine, l'expression de propos discriminatoires ou les appels à la violence doivent naturellement être sanctionnés. De tels propos nuisent en effet à l'essence même de notre État de droit et au débat républicain. Certains, dans l'hémicycle ou sur les bancs des ministres, en ont déjà été la cible. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'association Point de contact, reconnue pour son expertise dans la lutte contre les contenus pédopornographiques et terroristes. Cette association avait été présentée par le général de gendarmerie Watin-Augouard, fondateur du forum international de cybercriminalité, qui se tient tous les ans à Lille. Créée en 1998, Point de contact est une plateforme de signalement de contenus illicites et haineux à destination du grand public. Après avoir trié et qualifié juridiquement les contenus signalés, cette association permet de de transmettre à la plateforme Pharos du ministère de l'intérieur les alertes repérées pour que les autorités puissent ouvrir des enquêtes et engager d'éventuelles poursuites judiciaires.

de nombreux professionnels de la modération de contenus demandent que leur profession soit reconnue par la médecine du travail comme étant de grande pénibilité. Monsieur le secrétaire d'État, que pensez-vous de cette demande légitime ? Il faut aider ces structures, surchargées et en sous-effectifs, qui manquent de moyens. Car elles peuvent faire beaucoup dans cette lutte contre la haine.

En effet, préserver la liberté d'expression, lutter contre les contenus haineux sans censurer : il est bien difficile de cerner cette limite par la loi dans un monde complexe, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État. Nous devons protéger à tout prix cette liberté d'expression qui est garantie par la Constitution et qui pourtant recule partout en France. Je le dis fermement : notre liberté d'expression n'est pas négociable. Mais la liberté d'expression n'est pas la seule valeur de notre société : il y a aussi le respect, la décence, le bien commun. Nous devons aussi refuser et combattre cette augmentation et cette banalisation de la violence, décuplées par la puissance des réseaux sociaux qui, parfois, attisent et prêchent la haine. Nous devons aussi nous pencher sur les raisons de cette augmentation de la violence. Il y a aujourd'hui un problème d'éducation à cette liberté d'expression, à ses excès, mais aussi un vrai problème moral. Cette liberté d'expression n'est pas toujours bien comprise et bascule parfois dans la calomnie, l'injure, et produit ainsi de la violence. La liberté d'expression, c'est la contradiction, le débat, la recherche de la vérité. À l'époque des attentats de 2015, le philosophe Régis Debray avait une formule que je trouve intéressante : « Le désert des valeurs fait sortir les couteaux. »

je suis opposé à ce que les GAFA régulent notre liberté d'expression. Ne créons pas une police de la pensée. J'ajoute que la notion de « contenu haineux » n'est pas définissable et ne peut faire l'objet d'aucune définition juridique. Néanmoins, il me semble qu'il y a un vrai travail à faire en amont pour éduquer à l'esprit critique, à la raison, au débat dans le respect : on combat un adversaire non pas en le bâillonnement juridiquement, mais avec des arguments. Il faudrait pouvoir faire davantage de prévention et d'éducation sur une utilisation civique et responsable des réseaux sociaux.

monsieur le secrétaire d'État, je remercie le Gouvernement et l'ensemble de nos collègues de leurs contributions, de leurs analyses et de leurs propositions sur un sujet qui nourrit, à juste titre, beaucoup de débats en France, en Europe et dans le monde. Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, puis Instagram, Snapchat et, plus récemment, TikTok, tous rencontrent un succès assez phénoménal auprès de ceux qui ont accès à internet et aux smartphones. Si ces publications, ces, ces rencontrent un grand succès, c'est qu'ils répondent à des aspirations profondes : s'exprimer, communiquer, partager. Les réseaux sociaux ont bouleversé nos vies, le journal de vingt heures a été remplacé pour beaucoup par un fil d'actualité, l'article de presse, l'éditorial a été balayé par un, le le coup de fil à un ami s'est transformé en une accumulation de notifications et d'échanges de messages. On peut le regretter, on peut l'approuver, on peut le critiquer, mais, aussi vrai que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest, c'est un fait qui fait partie de nos vies et nous ne reviendrons pas en arrière. et nous sommes d'accord pour l'affirmer -une écrasante majorité utilise les réseaux sociaux de manière bienveillante, certains s'en servent pour développer des théories fumeuses pour déverser leur haine et pour insulter l'intelligence collective. Sous couvert de la liberté d'expression, ils mettent en danger la liberté, la vraie, celle des idées, celle des arguments, du débat, celle qui permet à une société de s'additionner et de progresser. Au final, ils nous interrogent et nous mettent devant nos responsabilités sur un enjeu essentiel, celui du vivre ensemble. La question qui nous est posée est celle-ci : comment trouver les moyens de réguler les réseaux sociaux ? Chaque Française, chaque Français, dans sa vie publique, doit, partout et chaque fois, prouver qui il est, assumer son identité, justifier de sa situation, d'un lieu d'habitation, montrer son visage. Partout et chaque fois, sauf sur internet et sur les réseaux sociaux ! Les Facebook, Google et Twitter sont trop contents d'accumuler, sans aucun contrôle, les profils, synonymes pour eux d'autant de pub'et de données à revendre. Il faut en finir avec le règne du pseudo-anonymat C'est la responsabilité individuelle qui crée les conditions du vivre ensemble. C'est l'anonymat qui crée l'irresponsabilité qui engendre, pour beaucoup, les débordements, les mises en cause et les insultes qui gangrènent les réseaux sociaux. La presse, la télévision, l'ensemble des médias sont responsables devant la loi des contenus qu'ils publient. Pourquoi en irait-il autrement des réseaux sociaux ? La même loi doit s'appliquer à tous les éditeurs de contenu. Les algorithmes de Google et de Facebook sont assez puissants pour connaître la marque des chaussures que nous portons, les lieux que nous fréquentons et les personnes que nous avons croisées récemment. Mais les mêmes algorithmes ne sont pas en mesure de bloquer les profils suspects, d'empêcher les appels à la haine et de casser les groupes de farfelus ou de dangereux qui se réunissent : mensonge, triple mensonge

pays d'Europe ont pris des mesures, qui ont en partie donné des résultats. En France, un pas avait été fait avec la loi Avia, dont les principaux articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Le législateur, le Gouvernement et les instances européennes doivent être à l'initiative d'un nouveau cadre qui contraindra les réseaux sociaux à lever l'anonymat et leur fera assumer leur responsabilité devant la loi.

loi doit être la même. » J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au retour de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.